Madame la présidente,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

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, comme à l'accoutumée, ma collègue Sophie Taillé-Polian et moi-même allons présenter, à deux voix, les crédits demandés par le Gouvernement pour Malgré des divergences, nous pouvons, dans certains cas, dresser des constats communs. En premier lieu, nous ne pouvons que nous féliciter de la hausse substantielle des crédits

Cette augmentation est d'autant plus nécessaire que la situation sur le marché du travail s'est brutalement dégradée. Pour ne donner qu'un chiffre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a déjà progressé de près de 10 %.

Les prévisions, déjà pessimistes, que nous présentons dans notre rapport ont elles-mêmes été établies avant la décision du second confinement ... Une certitude, cependant : les ajustements à ces chocs sur le marché du travail touchent en premier lieu les jeunes et les salariés les plus précaires.

Pour faire face à la crise, la mission « Plan de relance » alloue près de 10 milliards d'euros supplémentaires à la politique de l'emploi. Ces crédits renforceront des dispositifs existants et d'ores et déjà financés par la présente comme les parcours emploi compétences et la garantie jeunes. Ce choix est certainement le bon, car l'heure n'était pas à l'improvisation de mesures nouvelles dans la précipitation le principal enjeu est d'être en mesure de déployer les actions le plus rapidement et le plus puissamment possible. J'observe toutefois que, sur le strict plan de la lisibilité budgétaire, la situation n'est pas vraiment optimale. Prenons l'exemple de l'activité partielle alors que le dispositif de droit commun relevait de la mission « Travail et emploi », les 21 milliards d'euros débloqués au titre des lois de finances rectificatives pour 2020 ont été retracés sur un programme de la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire 2021, aucun euro n'est inscrit sur ce programme, puisque le dispositif sera financé sur une troisième mission- « Plan de relance Cette architecture ne permet pas aux parlementaires de connaître aisément et avec précision l'effort budgétaire que le Gouvernement entend consacrer à la politique de l'emploi, politique cruciale s'il en est pour l'année qui vient.

Sur le fond des politiques menées, la stratégie, sensiblement la même qu'au cours des années précédentes, me paraît aller dans le bon sens : concentrer les moyens sur les publics les plus fragiles grâce à des dispositifs ciblés

pour la deuxième année consécutive, que les crédits alloués au secteur de l'insertion par l'activité économique, qui emploie des personnes rencontrant des difficultés particulièrement fortes d'accès au marché du travail, dépassent le milliard d'euros. Les crédits mobilisés en faveur des travailleurs en situation de handicap au titre des aides au poste dans les entreprises adaptées progressent également. On relève aussi une augmentation des moyens alloués au dispositif des emplois francs,

En tout état de cause, les publics concernés par ces dispositifs sont frappés de plein fouet par la crise. Plus préoccupant encore, l'expérience des crises passées suggère que ces catégories ne bénéficieront pas spontanément des effets de la reprise, lorsqu'elle aura lieu

est, dans l'ensemble, un budget sérieux et nécessaire. C'est pourquoi la commission des finances recommande au Sénat d'adopter les crédits de la mission « Travail et emploi ».

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, mon analyse du budget qui nous est proposé pour la mission « Travail et emploi »

sens, il ne faut pas en exagérer la portée : elle est simplement conforme à la trajectoire prévue par la loi de programmation des finances publiques votée en 2018, qui inscrit le ministère du travail et le nombre de ses fonctionnaires dans une trajectoire de diminution-

On ne soulignera jamais assez que cette mesure revient,, à faire supporter par les chômeurs eux-mêmes le coût du service public de l'emploi. Ainsi, la nécessité d'améliorer les comptes de l'assurance chômage, déjà lourdement affectés par la crise et la prise en charge du chômage partiel, risque, demain, de

La forte dégradation attendue de la situation sur le marché du travail et ses conséquences sociales de long terme appelleraient, à l'inverse, une augmentation pérenne et structurelle des effectifs. De même, on peut s'interroger sur l'urgence qu'il y a à poursuivre, un peu à marche forcée, la réforme de l'organisation territoriale de l'État (OTE), qui concerne tout particulièrement les ministères sociaux. Pour ma part, je crains que cette réforme n'entraîne une certaine désorganisation, à l'heure où les services devraient être totalement tournés vers la gestion des conséquences de la crise. Il y a, certes, des aspects positifs dans ce budget, comme les moyens conséquents prévus en faveur de l'inclusion dans l'emploi des publics les plus fragiles, notamment dans le secteur de l'insertion par l'activité économique. Mais certaines questions se posent,

les plus fragiles sur une logique d'insertion par l'activité, je vous indique que la commission des affaires sociales a émis sur les crédits un avis favorable. Pour autant, je ne cache pas avoir ressenti un certain étonnement en découvrant ce budget. En effet, les crédits demandés augmentent légèrement par rapport à la loi de finances initiale pour 2020, ils restent inférieurs aux crédits consommés cette année, compte tenu des quatre lois de finances rectificatives intervenues jusqu'à présent. Surtout, la mission que nous examinons ce matin ne comporte aucune mesure nouvelle et s'inscrit dans la droite ligne des budgets des années précédentes- s'agissant de ce que nous avons approuvé, mais aussi de ce que nous avons critiqué. On pourrait presque croire que la situation de l'emploi dans notre pays n'a guère changé en un an, et que la dynamique de baisse du chômage que nous observions à la fin de 2019 s'est poursuivie ... Or, chacun le sait, la crise sanitaire a entraîné une remontée spectaculaire du taux de chômage, qui ne devrait pas retrouver son niveau du premier trimestre 2020 avant plusieurs années.

Elle ne paraît pas toujours justifiée et tend à donner une image quelque peu inexacte de la politique menée. Ainsi, le plan de relance finance en partie l'extension de dispositifs financés à titre principal par la mission « Travail et emploi il est difficile de concevoir en quoi l'accompagnement de 100 000 jeunes par la garantie jeunes relèverait de la politique normale de l'emploi, mais que 50 000 jeunes supplémentaires seraient, par ailleurs, accompagnés dans le cadre du plan de relance du plan d'investissement dans les compétences (PIC), correspondant en fait au financement de dispositifs déjà pérennisés, comme la garantie jeunes, ainsi qu'à une enveloppe attribuée au Gouvernement sans que le Parlement et les partenaires sociaux en connaissent l'utilisation exacte. La Cour des comptes a critiqué ce manque de clarté, alors que les crédits que nous votons à ce titre sont chaque année sous-consommés. Comme les années précédentes, l'État bénéficierait d'un fonds de concours de France compétences. La Cour des comptes a eu l'occasion d'émettre des doutes sur la régularité de ce fonds de concours dont l'État fixe lui-même le montant. Ce prélèvement de 1,6 milliard d'euros sur les ressources de France compétences s'accompagne, en sens inverse, d'une subvention exceptionnelle de 750 millions d'euros. Ainsi, le Gouvernement parvient à gonfler à la fois le PIC et le plan de relance, au détriment de la lisibilité pour le Parlement. Je remarque en outre que le Gouvernement tire les conséquences du déséquilibre créé par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Tous, dans cet hémicycle, nous craignions qu'il ne conduise à faire du financement de l'apprentissage une variable d'ajustement du budget de France compétences. Une étude d'impact plus solide aurait sans doute été utile

Dans cette période difficile, le ministère du travail joue un rôle fondamental. Je salue l'engagement des agents du ministère et de ses opérateurs, très mobilisés sur le terrain.

les crédits de la mission « Travail et emploi » constituent le budget socle du ministère, en augmentation de 400 millions d'euros conformément aux trajectoires prévues avant la crise. D'autre part, les crédits exceptionnels de la mission « Plan de relance » s'ajoutent à cet effort : sur les 22 milliards d'euros de France Relance, 10 milliards d'euros sont fléchés vers le ministère du travail pour renforcer son budget socle et l'efficacité de son action en faveur de la formation et de l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi. Au travers de ces crédits, on peut distinguer quatre priorités. Premièrement, protéger l'emploi. À cette fin, 7,6 milliards d'euros, dont 2,2 milliards d'euros financés par l'Unédic, permettent de créer un bouclier anti-licenciements, articulé autour de deux objectifs principaux : prendre en charge l'activité partielle et la formation des salariés pendant leur temps non travaillé et réarmer les entreprises pour qu'elles sortent de la crise plus compétitives, grâce à des salariés plus compétents. Dans ce cadre, 500 millions d'euros seront attribués au dispositif Transitions collectives, qui favorise les transitions professionnelles interbranches. Un appel à manifestation d'intérêt sera d'ailleurs lancé prochainement pour déployer ce dispositif auprès de bassins d'emplois pilotes. Deuxièmement, donner aux jeunes des solutions d'insertion. Pour ce faire, le ministère du travail pilote la plus grande partie des 6,7 milliards d'euros du plan « 1 jeune 1 solution » : 5,7 milliards d'euros, dont 3,6 milliards d'euros Ce plan comporte deux axes : le soutien à l'embauche, grâce aux primes exceptionnelles pour encourager les embauches de jeunes et les signatures de contrat en alternance ; le renforcement des dispositifs d'accompagnement et d'inclusion des jeunes. Au total, près de 300 000 places supplémentaires en accompagnement et inclusion sont prévues à destination des jeunes en garantie jeunes, en parcours contractualisé d'accompagnement adapté vers l'emploi et l'autonomie (Pacea)- en plus des places déjà prévues dans le budget socle - et en accompagnement intensif jeunes par Pôle emploi. Parce que les jeunes doivent être le coeur de notre attention durant cette crise, nous saluons l'importance des 100 millions d'euros supplémentaires qui renforceront le budget des missions locales. Mais il nous a paru important de déposer à cet égard deux amendements.

Le second vise à étendre, sur arrêté ministériel, le bénéfice de la protection sociale et de la rémunération attachées au statut de stagiaire de la formation professionnelle aux jeunes bénéficiaires des dispositifs d'accompagnement, d'insertion professionnelle, de stage Le tout dans le cadre d'un programme national destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de personnes en recherche d'emploi. Troisièmement, développer les dispositifs d'insertion sur mesure,

Alors que 20 000 parcours emploi compétences supplémentaires étaient prévus dans le budget socle, il a été décidé d'en ajouter 60 000 à destination des jeunes. Par ailleurs, 204 millions d'euros sont alloués aux dispositifs d'insertion par l'activité économique, dont 62 millions d'euros issus du plan de relance. Le budget alloué aux entreprises adaptées pour les personnes en situation de handicap augmente de 23 millions d'euros et favorise les passerelles vers les entreprises de droit commun. L'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » bénéficie, quant à elle, de 11 millions d'euros supplémentaires pour le financement de sa deuxième phase.

départementaux. Tous ces leviers sont actionnés pour prévenir les risques de basculement de nos concitoyens dans la pauvreté. Mais ils ne peuvent s'envisager qu'avec le déploiement d'un effort substantiel de formation, tout au long de la vie professionnelle. Telle est la quatrième priorité le plan d'investissement dans les compétences bénéficie d'un nouvel engagement de 3,3 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent, dans le cadre du plan de relance, près de 1,7 milliard d'euros destinés au financement des formations aux métiers d'avenir ou en tension. Comme de nombreux services, l'offre de formation continue se digitalise. Aussi l'État engage-t-il 500 millions d'euros pour aider à sa numérisation. Mes chers collègues, l'État est pleinement mobilisé Bien que très attentif à la maîtrise des dépenses publiques, il donne, au travers de ces budgets, de solides garanties et des moyens sans précédent pour que chacun puisse accéder à l'emploi ou s'y maintenir et que chaque entreprise ait les compétences nécessaires aux métiers de demain.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire, donc sociale et économique, que nous traversons est inédite et, à bien des égards, historique. Alors que plus de 400 000 emplois ont été créés en 2019, cette dynamique a été stoppée net par la covid-19. Les chiffres sont sans appel : avec 5,7 millions de personnes en recherche d'emploi en France métropolitaine, le taux de chômage s'est envolé à 9 % au troisième trimestre

Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle engendre des destructions durables d'emploi. Dans ce contexte particulièrement difficile, je salue l'augmentation des crédits de la mission « Travail et emploi », qui s'élèveront l'année prochaine à 13,4 milliards d'euros-

Vous prévoyez également de doubler le nombre de bénéficiaires de la garantie jeunes, ce qui porterait leur nombre à 200 000 en 2021. Dans ce climat singulièrement délétère pour l'emploi, il est impératif de prêter une attention toute particulière aux jeunes, mais également aux plus fragiles et aux plus précaires. Aussi accueillons-nous très favorablement le renforcement du dispositif « territoires zéro chômeur de longue durée ». Doté initialement de 22,61 millions d'euros, il bénéficiera finalement d'une enveloppe supplémentaire de 6 millions d'euros votée par l'Assemblée nationale. Cet effort permettra d'accompagner la montée en charge de l'expérimentation, étendue à cinquante nouveaux territoires au moins, dont Bordeaux et Castillon-la-Bataille, en Gironde.

Dans le projet de loi de finances initial, l'État prévoyait, pour la troisième année consécutive, de se désengager totalement du budget de fonctionnement de ces maisons, qui pourtant garantissent un socle de services universels de proximité et remédient aux angles morts des politiques publiques. et souples, ces structures peuvent être mobilisées rapidement et efficacement pour lutter contre les freins à l'emploi. Elles interviennent d'ailleurs dans des domaines qui ne sont pas toujours couverts par les services publics de l'emploi. L'État peut s'appuyer sur elles pour déployer des politiques prioritaires, comme la clause d'insertion sociale, qui présente un taux d'insertion que peu de structures peuvent aujourd'hui

Depuis le 2 mars, 67 000 emplois ont été supprimés ; malheureusement, nous savons que ce n'est pas terminé. Nous pensons à tous ces petits commerçants qui ne se remettront pas de ce deuxième confinement, et qui emploient parfois une ou deux personnes, ou encore aux

Alors qu'il faudrait renforcer le service public pour amortir la crise, le Gouvernement diminue les crédits destinés à l'amélioration de l'efficacité de Pôle emploi. Il diminue les crédits pour la santé et la sécurité au travail. Il diminue les crédits pour le dialogue social et la démocratie sociale de 18 %, alors qu'il aurait fallu les privilégier, surtout en cette période. Alors qu'il faudrait anticiper les plans de licenciements, le Gouvernement diminue les crédits pour l'anticipation et l'accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l'emploi de 34 % par rapport à 2020. Enfin, alors qu'il faudrait renforcer les services d'accompagnement des privés d'emploi, le Gouvernement diminue les crédits pour les personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et de développement de l'emploi. La politique à contresens du Gouvernement nous dirige droit dans le mur. de la réforme de l'assurance chômage, le Conseil d'État a retoqué la réforme Pénicaud, qui prévoyait de durcir les critères d'accès et l'annulation des droits rechargeables. Cette décision est une victoire pour les précaires. C'est maintenant la réforme de l'assurance chômage qui doit être supprimée dans son intégralité, comme le demande l'ensemble des organisations syndicales.

Année après année, ces coupes dans les effectifs fragilisent les missions assurées notamment par l'inspection du travail et les maisons de l'emploi.

Le Gouvernement agit dans l'urgence et tente de colmater les brèches. Il annonce régulièrement de nouvelles dépenses, parfois en milliards d'euros, sans malheureusement toujours s'inquiéter de leur approbation préalable par le Parlement.

Nous espérons sincèrement que ce découpage ne remettra pas en cause l'ambition des politiques menées. Sur le fond, la stratégie est finalement la même que les années précédentes, les objectifs étant de concentrer les moyens sur les publics les plus fragiles grâce à des dispositifs ciblés

par l'activité économique (IAE) et au renforcement du plan d'investissement dans les compétences (PIC). L'IAE contribue au développement économique des territoires par la création d'activités économiques ancrées localement. Elle constitue une réponse structurelle à l'objectif d'insertion professionnelle des personnes très éloignées du marché du travail, qui ne bénéficient pas spontanément de la reprise économique et pour lesquelles la seule formation professionnelle ne constitue pas une réponse adaptée. Nous notons aussi l'instauration de dispositifs de prime à l'embauche et la mobilisation accrue des dispositifs de contrats aidés. La prime à l'embauche facilite l'embauche immédiate pour un grand nombre de publics- apprentis, jeunes et travailleurs handicapés. Quant à la mobilisation accrue des dispositifs de contrats aidés, nous n'avons cessé d'en défendre la pertinence. Certains de nos concitoyens sont plus fragiles du fait d'une expérience de vie malheureuse ou d'un accident ; ils ont besoin d'un coup de pouce, d'une main tendue pour retrouver un lien avec le monde du travail : tel est le rôle des contrats aidés, surtout en période de crise sociale. Ils permettent d'inclure dans l'emploi des publics qui en sont éloignés et renforcent notre tissu associatif et nos collectivités. Par ailleurs, nous regrettons

que je suis fermement opposé à cette politique du chiffre : tous les jeunes doivent trouver une porte ouverte dans le service public, à plus forte raison quand toutes les autres leur sont fermées. Le service public s'adresse à tous, plus particulièrement à ceux qui en ont le plus besoin. La mission « Travail et emploi » est marquée par la montée en puissance des dispositifs d'insertion, dont la formation professionnelle est un volet majeur. En tant qu'orateur de mon groupe lors de l'examen du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, j'avais salué certains des objectifs tout en m'inquiétant de leur mise en oeuvre.

de la formation professionnelle. Leur engagement sur ces sujets est exemplaire ; nous regrettons que le plan de relance ne les laisse trop à l'écart, car elles sont l'échelon le plus pertinent pour jouer un rôle de pilotage de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi.

des CDI crée une dynamique très positive pour eux-mêmes et pour leur territoire. Ce projet est issu de l'expérience d'acteurs de terrain et du tissu associatif. Il est la preuve que nous devons permettre à nos collectivités locales et aux corps intermédiaires d'être forces de proposition

d'entrer dans les prochains mois dans une crise économique et sociale très forte. Le vent va souffler, car à la crise sanitaire risque de succéder une crise sociale-

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le monde est confronté à une crise sanitaire et économique sans précédent dont on ne mesure pas encore l'ampleur. Il est d'autant plus difficile de faire des projections que la situation sanitaire reste incertaine. Selon les prévisions de l'Insee, le PIB de la France pourrait baisser de 9 % en 2020, et le rebond serait, non plus de 8 %, mais de 6 % en 2021. Le recours massif au dispositif exceptionnel d'activité partielle a certes permis de contenir les licenciements, mais il ne suffira pas à empêcher une forte hausse du chômage dans la période qui s'ouvre. Plus de 35 000 suppressions de postes ont été annoncées depuis septembre, et les experts alertent sur une probable explosion des plans sociaux et des faillites l'an prochain. Au troisième trimestre 2020, le taux de chômage a déjà bondi de 1,9 point, touchant plus de 2,7 millions de Français. Alors que des dispositifs comme le chômage partiel ou la prime d'activité permettent de limiter la perte de pouvoir d'achat des salariés modestes, il y a à l'évidence une urgence sociale : il urgence sociale : il faut venir en aide aux Français qui, avant la crise, évoluaient dans une zone grise, cumulant des petits boulots, et qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi, fragilisés de surcroît par la réforme de l'assurance chômage. Le 25 novembre dernier, le Conseil d'État rendait une décision faisant suite à l'examen de différents décrets relatifs à la réforme de l'assurance chômage promue jusqu'à l'entêtement par le Gouvernement.

Cette disposition retenue unilatéralement par le Gouvernement vient d'être censurée par le Conseil d'État au motif d'une atteinte au principe d'égalité. Depuis plus d'un an, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain n'a cessé de dénoncer les effets dévastateurs de cette réforme profondément injuste, dont l'objectif inavoué est de réduire le nombre de demandeurs d'emploi éligibles à une inscription tout en diminuant l'indemnisation de nombreux autres chômeurs, et alors que les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire aggravent encore les effets attendus de cette réforme, selon la dernière étude d'impact de l'Unédic. Le Conseil d'État vous ayant infligé un nouveau camouflet, nous vous invitons encore et toujours à reprendre le chemin de la démocratie sociale et de la négociation. La première suspension de la réforme était bienvenue, mais il aurait fallu qu'elle soit totale, qu'elle prévoie le rechargement des droits et qu'elle concerne également les personnes ayant perdu leur emploi entre novembre 2019 et août 2020.

Avec la crise de la covid-19, plus de 1 million d'entre eux ont perdu leur source de revenus. Très juste ! Ils sont de surcroît victimes des premiers effets de la réforme de l'assurance chômage. Le Président de la République paraissait avoir pris en compte la situation de ces travailleurs, si, de prime abord, les annonces de son Premier ministre ont semblé répondre aux attentes, elles se sont révélées décevantes. Une prime exceptionnelle de 900 euros pendant quatre mois, qui ne devrait bénéficier qu'à 300 000 personnes

J'en viens plus précisément aux crédits de la mission « Travail et emploi ». Nous prenons acte de leur augmentation, qui porte leur total à plus de 13 milliards

À l'image de mes collègues, je regrette cependant que l'éclatement du financement de la politique de l'emploi en 2021 entre les deux missions se fasse au détriment de la lisibilité budgétaire pour le Parlement. Comme l'an dernier, la principale hausse concerne le plan d'investissement dans les compétences. Nous vous retrouvons dans le soutien à la formation et dans le plan de relance en faveur de l'apprentissage.

de la formation professionnelle engagée par votre prédécesseur, madame la ministre. L'inspection générale des affaires sociales et l'inspection générale des finances estiment en effet dans le rapport publié en septembre qu'il manquerait 4,9 milliards d'euros pour la période 2020-2023. Il faut donc trouver des financements afin d'assurer la pérennité de cette réforme ; pourtant, votre projet de budget ne prévoit pas d'octroyer une subvention suffisante à France compétences. Autre source d'inquiétude : année après année, les coupes dans les effectifs fragilisent les missions assurées par le ministère du travail et les services déconcentrés, notamment l'inspection du travail, dont le rôle est pourtant essentiel pour garantir le respect des droits des salariés. L'État poursuit également son désengagement dans le financement de Pôle emploi, dont les subventions diminuent au moment même où les ressources de l'opérateur provenant d'une fraction des cotisations d'assurance chômage s'effondrent. Si Pôle emploi bénéficie, pour faire face à la forte hausse du nombre de demandeurs d'emploi, d'une enveloppe exceptionnelle dans le cadre du plan de relance, celle-ci est bien loin de compenser la baisse cumulée de ses subventions de fonctionnement depuis le PLF 2018. Au final, l'opérateur manque de visibilité, alors que la crise durable que nous traversons devrait plutôt inciter à proposer des accompagnements pérennes et renforcés. Pour finir, je souhaite à mon tour évoquer l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », que je connais bien. À Colombelles, dans mon département du Calvados, l'expérience menée depuis 2016 est très positive et concluante, de sorte que j'ai toujours été favorable à son extension. Bien qu'éloignée de la philosophie initiale de la démarche, et même si toutes les garanties que nous demandions n'ont pas été apportées, je suis satisfaite que le Parlement ait adopté il y a quelques jours la proposition de loi relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée

partenariale et territoriale dans la lutte contre le chômage. Elle met également en exergue la volonté des bénéficiaires de travailler, car, contrairement à certaines idées reçues, les personnes privées d'emploi ne se complaisent pas dans les allocations. Du reste, beaucoup ne sont plus indemnisées. Ce dispositif aura surtout permis de rendre visibles des personnes qui avaient totalement disparu des indicateurs du chômage. Dans les territoires zéro chômeur de longue durée, une amélioration des parcours de vie est à noter. L'essentiel des personnes que j'ai rencontrées considère ce dispositif comme une véritable chance : elles peuvent ainsi sortir de leur isolement social et se sentir de nouveau reconnues. L'entrée dans l'entreprise à but d'emploi en CDI leur permet de vivre leur quotidien plus sereinement

ont voté les mesures prises par le Gouvernement en faveur de l'emploi et de l'activité partielle. Toutefois, pour toutes les raisons évoquées, et surtout parce que la réforme de l'assurance chômage n'est toujours pas abrogée, ils prendront de nouveau leurs responsabilités en s'abstenant lors du vote des crédits de la mission « Travail et emploi

la mission « Travail et emploi » s'inscrit cette année dans un contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire. La deuxième vague de l'épidémie de covid-19 et les mesures sanitaires qui y sont liées ont déjà et auront encore des conséquences sur l'emploi qu'il nous faut anticiper pour en éviter les pires effets. Alors que les prévisions du taux de chômage à court terme se situent entre 9,8 % et 11 %, la France ne saurait se résigner à un chômage de masse et de longue durée. Il nous faut lutter contre cette fracture sociale qui s'aggrave chaque semaine. Or le budget 2021 ne semble pas suffisamment tourné vers cet objectif. Le chômage partiel en est le premier exemple. Si la prise en charge de l'activité partielle pendant le premier confinement a pu être absorbée grâce au pragmatisme des chefs d'entreprise, la deuxième vague de l'épidémie a changé la donne. Beaucoup redoutent désormais une onde de choc, qui requerra un accompagnement financier massif des entreprises, et des crédits pour former les nouveaux demandeurs d'emploi, notamment aux nouveaux métiers liés au numérique et à l'intelligence artificielle. de financer cet accompagnement ni dans cette mission ni dans la mission « Plan de relance », les crédits de cette dernière visant seulement à assurer le maintien d'une partie des salaires. À ce propos, la dégradation spectaculaire des comptes de l'Unédic, dont la dette devrait dépasser 65 milliards d'euros en 2020, est très largement due aux décisions de l'État en matière d'activité partielle. La question de la gestion de cette dette devra donc se poser ; il semblerait logique que l'État en prenne sa part. Notons également que les ressources de Pôle emploi sont fortement liées à celle de l'Unédic, avec un effet retard de deux ans. La dégradation des comptes de l'assurance chômage créera donc d'importantes difficultés de fonctionnement pour Pôle emploi dès 2022 et elle aura une répercussion sur les formations, pourtant si nécessaires pour l'avenir des emplois. La récession actuelle entraînera un afflux de demandeurs d'emploi vers les structures chargées de l'accompagnement et de la réinsertion professionnelle. Or le financement de la formation professionnelle a été mis à mal par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les OPCO, les branches professionnelles, les régions ne retrouvent pas les crédits utiles à l'accompagnement. Au déséquilibre financier qui en résulte s'ajoute désormais une baisse des recettes assises sur la masse salariale. Le scénario semble joué d'avance : les gros CFA et autres centres de formation vont bien s'en sortir, mais les plus petits auront besoin d'être refinancés. Encore une fois, ce sont les jeunes du monde rural qui seront pénalisés. Autre interrogation : le Gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs de prime à l'embauche pour un grand nombre de publics : apprentis, jeunes, travailleurs handicapés. Ces primes facilitent l'embauche immédiate, mais, ces dispositifs prenant fin en mars 2021, on peut légitimement s'interroger sur la rentrée 2021 : ces mêmes publics risquent alors de rencontrer des difficultés pour trouver un employeur. Les entreprises participent déjà à la formation la taxe d'apprentissage, l'alternance et la formation continue. Doivent-elles prendre toute la formation à leur charge ? Faire face au défi du chômage, c'est aussi veiller à ce que les travailleurs seniors ne soient pas exclus du marché de l'emploi. L'enjeu est moins d'allouer des exonérations incitatives qui ne fonctionnent pas que de faire de la psychologie pour que les chefs d'entreprise changent de regard et cessent de se séparer de cette main-d'oeuvre précieuse par des licenciements ou des ruptures conventionnelles lors des dernières années de carrière. La crise risque en effet d'avoir des conséquences lourdes pour les seniors. Au cours des trois dernières années, la progression des inscriptions de seniors à Pôle emploi a été de 12 % par an, soit deux fois supérieure à celle des jeunes. De plus, les seniors restent inscrits au chômage trois fois plus longtemps. Je rappelle qu'en juillet 2019, dans un rapport, la Cour des comptes avait constaté l'absence de stratégie nationale en matière d'emploi des seniors. Or rien n'a changé depuis. Enfin, la crise sanitaire a bouleversé nos méthodes de travail, entraînant un recours massif au télétravail sans pour autant faire disparaître les risques professionnels. Aussi, je regrette la diminution des crédits de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail alors que les besoins en prévention sont très importants, que ce soit pour la prise en charge des troubles musculo-squelettiques, qui ne figurent pas dans le projet annuel de performance, pour celle des risques psychosociaux, qui augmentent, ou encore pour l'accompagnement des très petites entreprises dans l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels.

comme toutes les missions que nous avons examinées cette année, la mission « Travail et emploi » est placée sous le signe de la covid. La crise, qui a d'abord mis à mal notre système de santé, a ensuite frappé notre économie de plein fouet. Pourtant, de nombreux indicateurs laissent penser que nous n'avons pas encore constaté toute l'ampleur des dégâts ; cela vaut tout particulièrement pour le marché du travail, qui a bénéficié d'amortisseurs très puissants, notamment grâce au dispositif Une vague de faillites et de licenciements pourrait ainsi frapper le pays de façon décalée, mais non moins violente. Alors que le taux de chômage atteint déjà 9 %, il est à craindre que la situation continue de se dégrader. C'est dans ce contexte très difficile que nous examinons les crédits consacrés à cette mission. Ses programmes s'inscrivent dans une logique contracyclique les crédits alloués sont appelés à augmenter quand la situation se détériore et à diminuer lorsqu'elle s'améliore. C'est pour cela que le groupe Les Indépendants a soutenu au cours des dernières années la baisse courageuse des crédits de la mission.

Il ne s'agit pas d'inverser la tendance, mais de suivre la même logique : agir de façon contracyclique. La hausse des crédits correspond pour l'essentiel à des mesures plus conjoncturelles que structurelles, en visant en priorité le retour à l'emploi et en articulant solidarité et efficacité. En temps de crise comme en temps normal, la meilleure politique sociale consiste à permettre à chacun de trouver l'emploi qui lui convient. Plusieurs des mesures proposées me paraissent ainsi aller dans le bon sens. Je pense tout d'abord au rétablissement des contrats aidés dans le secteur marchand. Comme l'a rappelé le rapporteur spécial, subventionner l'emploi ne saurait constituer l'alpha et l'oméga d'une politique économique, dont l'objectif doit être de dynamiser le marché du travail. C'est pourquoi notre groupe avait approuvé la suppression de ce dispositif.

À cet égard, le cas des outre-mer s'avère intéressant. En effet, les emplois aidés devenus parcours emploi compétences ont toujours été plus dotés dans les territoires ultramarins qu'en métropole, compte tenu de la situation plus dégradée du marché du travail. Or ces

La crise actuelle nous a, à bien des égards, redonné le goût du terrain. Nous reprenons conscience que c'est en nous appuyant sur les acteurs locaux et les structures de proximité que nous parvenons globalement aux meilleurs résultats. C'est pourquoi je partage l'analyse des deux rapporteurs spéciaux sur la nécessité de renforcer les moyens alloués aux maisons de l'emploi. Le Gouvernement devrait sur ce point écouter les propositions de la commission des finances, car elles relaient les demandes du terrain. De même, je partage les regrets formulés sur la qualité d'exécution du plan d'investissement dans les compétences, dont les crédits avoisineront les 3,4 milliards d'euros où nous déployons des moyens faramineux pour déclencher un électrochoc sur notre économie, il n'est pas acceptable de constater des pertes en ligne ou du retard au démarrage. Il y va de l'efficacité de la relance. Plus fondamentalement, il y va aussi de la confiance que les Français accorderont à la parole politique. En effet, l'on peut bien annoncer et voter tous les plans de relance que l'on veut ; si nos concitoyens n'en voient pas la couleur sur le terrain, alors c'est la parole politique qui perd en crédit. La défiance ne doit pas entamer les efforts que nous allons consentir collectivement. Il est important que nous ne laissions pas s'installer le sentiment, selon lequel certains profitent indûment du système.

alors que la crise sanitaire démultiplie les crises économique et sociale, nous avions besoin de politiques du travail et de l'emploi renouvelées et justes. Or dans l'ensemble, hormis l'impact du plan de relance, qui brouille d'ailleurs la lisibilité de la politique budgétaire, les mêmes politiques se poursuivent. Cette mission n'enregistre guère de mesures nouvelles et ses crédits évoluent sous l'effet des décisions antérieures, la trajectoire retenue depuis 2017 Plus qu'une continuité de trajectoire, la situation exige une rupture pour faire face à la dégradation profonde et brutale du marché de l'emploi et à la crise sociale. Le chômage explose, alors que le choc est encore à venir dans les secteurs touchés de plein fouet par la crise. Au niveau national, il dépasse 9 % de la population active. Rien que dans le Rhône, il progresse de plus de 10 % au troisième trimestre de cette année 2020 par rapport à celui de 2019. Dans la seule métropole lyonnaise, près de 2 000 emplois sont désormais chez Renault Trucks. Ces destructions d'emplois ne sont pas toutes dues à la crise sanitaire. De grands groupes profitent du contexte pour délocaliser et monter des plans sociaux.

a été patiemment reconduite depuis le début du quinquennat, mais elle est encore plus injustifiable, alors que la situation s'est dégradée bien au-delà de l'impact mécanique de la crise. À l'issue du plan de relance, entre destructions et créations d'emplois, les données indiquent une augmentation de 200 000 chômeurs par rapport à l'avant-crise et de nombreux chômeurs basculeront dans le chômage de longue durée. Félicitons-nous, dès lors, de retrouver au moins les crédits de l'extension du dispositif « territoires zéro chômeur de longue durée » adopté récemment et soutenu par le groupe

Il faut renforcer les politiques d'insertion et de soutien au travail, car la crise ne se réduit pas à un accident conjoncturel. L'explosion du télétravail, entre autres bouleversements, oblige à contester la baisse des budgets de la santé au travail comme des moyens de contrôle du ministère. Nous présenterons également des amendements

Si la mission consacre à juste titre un soutien accru au secteur de l'insertion par l'activité économique, il conviendra de veiller au maillage territorial. Nous approuvons le retour des emplois aidés, hélas pointé comme exceptionnel. Le Gouvernement maintient en effet son analyse, selon laquelle il s'agit seulement d'un traitement statistique du chômage qu'il stoppera dès la reprise.

Enfin, nous souhaitons que le coût de la politique gouvernementale de recours massif à l'activité partielle, politique bienvenue, soit isolé et pris en charge en partie par l'État, pour ne pas justifier à l'avenir des mesures de réductions des droits, comme dans la réforme de l'assurance chômage dont nous continuons

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le fort recul de l'activité économique mondiale en raison de la crise sanitaire se traduit par la fermeture de nombreuses entreprises et par une forte augmentation du chômage. Ainsi, selon la Dares, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, plus de 650 plans de sauvegarde de l'emploi ont été lancés en France. Dans les entreprises plus petites, de moins de dix salariés, on compte plus de 4 000 licenciements collectifs cumulés depuis mars. Les conséquences des plans sociaux annoncés ne sont pas encore visibles sur la courbe du chômage. Les entrées en formation et les dispositifs d'aides publiques permettent d'amortir l'impact de la crise sanitaire.

Les différents instituts de prévision retiennent, avec les précautions nécessaires dans un contexte inédit, l'hypothèse d'un taux de chômage compris entre 9,8 % et 11 % dans les prochains mois. Certes, la crise est conjoncturelle, mais elle est aggravée par l'absence de réformes structurelles. Les décisions prises actuellement sont des solutions d'urgence et de court terme. Dans ce contexte, l'augmentation de 400 millions d'euros des crédits de la mission « Travail et emploi », soit une hausse de 3 %, peut sembler insuffisante. La politique de l'emploi est surtout soutenue par la mission « Plan de relance », avec près de 10 milliards d'euros qui viendront en grande partie abonder des dispositifs déjà prévus par la mission. mission. L'éclatement du financement de la politique de l'emploi sur ces deux missions pose un réel problème de lisibilité budgétaire. Des questions surgissent également sur la pérennité des ressources pour les budgets à venir. En ce qui concerne l'apprentissage, nous ne pouvons que nous réjouir de l'augmentation du nombre de contrats d'apprentissage, qui jusqu'à la crise sanitaire a connu une forte dynamique, puisque la progression a été de 16 % par rapport à l'année précédente.

d'apprentis (CFA) qui dépendent de secteurs fortement atteints par la crise sanitaire pourraient rencontrer de sérieuses difficultés financières. Dans ce contexte, la stabilité des crédits reversés aux régions pour le financement de l'investissement et du fonctionnement des CFA questionne.

Toutefois, les entreprises adaptées ont été durement touchées par les conséquences de la crise sanitaire, avec une baisse de chiffre d'affaires estimée à 25 %. Il convient donc de les soutenir dans cette période difficile. Malgré nos inquiétudes, nous approuvons la mission « Travail et emploi » et les actions engagées par le Gouvernement dans le cadre du plan de relance. Néanmoins, nous restons inquiets du manque de réformes structurelles dans le domaine de l'emploi et, surtout, de l'application de la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle.

Madame la ministre,